aux chaînes parlementaires, au Conseil constitutionnel et à la Cour de justice de la République, tant que celle-ci existera. Parmi les traits saillants de ce budget, on observe

Ce gel sur neuf exercices consécutifs, si l'on prend en compte l'inflation, représente l'équivalent d'une année de dotation

La présidence et les assemblées sont engagées dans d'importants projets immobiliers, inscrits dans un cadre pluriannuel. Il s'agit d'un sujet majeur, parce que cela

notamment au bâtiment de l'Alma, même s'il n'est pas idiot de prévoir une maîtrise d'ouvrage globale. Pour financer tous les projets, ces institutions, notamment les assemblées, font appel à des prélèvements sur leurs réserves-

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une hausse de 3,6 % des crédits de la mission « Conseil et contrôle de l'État », qui sera ainsi dotée de 705 millions d'euros. Cette hausse, non prévue par la programmation triennale, bénéficie essentiellement au programme « Conseil d'État et autres juridictions administratives », qui voit ses crédits progresser de 19,5 millions d'euros. Cette augmentation devrait notamment contribuer à la création de 93 emplois, dont 59 postes au profit de la Cour nationale du droit d'asile Les moyens alloués à cette juridiction progresseront ainsi de plus de 20 % pour atteindre 67,5 millions d'euros, soit un niveau inédit jusqu'à présent. Monsieur le ministre, cette hausse n'a pas été anticipée par la loi de programmation des finances publiques et se traduit par un dépassement de plus de 5 % du plafond de la programmation triennale. comment ne pas y être favorable, alors que le contentieux de l'asile s'est littéralement envolé au cours des deux dernières années ? Je m'arrêterai un instant sur les chiffres : le nombre d'affaires à traiter,

C'est ce que fait ce budget pour 2020 et je m'en félicite : les 59 nouveaux emplois prévus pour 2020 devraient porter la capacité de jugement de la CNDA à près de 90 000 affaires par an en 2021. Les effectifs de la CNDA seront donc, à terme, suffisants chaque année pour absorber les nouvelles affaires, si tant est que leur nombre se stabilise dans les années à venir. Par ailleurs, cette année encore, cette augmentation laisse craindre un effet d'éviction aux dépens des autres juridictions administratives qui sont, elles aussi, confrontées à une hausse de leur contentieux, principalement imputable au contentieux des étrangers. Ce type très spécifique de contentieux représente plus de 98 000 nouvelles affaires en 2018, soit plus du tiers des flux dans les juridictions administratives et près de 50 % des flux dans les cours administratives d'appel. Il y a fort à craindre que cette dynamique finisse par peser sur les délais de jugement des juridictions administratives. Dans ce contexte, je note que le Premier ministre a confié au Conseil d'État le soin de réfléchir à une réforme du droit des étrangers pour simplifier les procédures liées à ce contentieux. Monsieur le ministre, sauriez-vous nous dire où en est cette réflexion et quelles sont les pistes de réforme étudiées ? Je serai plus bref sur les crédits des autres programmes, qui sont quasiment stables par rapport à 2019. Le budget du Conseil économique, social et environnemental (CESE) bénéficiera d'une augmentation de 4,2 millions d'euros, pour permettre l'organisation d'une deuxième convention citoyenne le savez, mes chers collègues, en réponse à la crise des « gilets jaunes », le Président de la République a confié au CESE l'organisation d'une convention citoyenne pour le climat, dont les membres sont chargés de formuler des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici à 2030. Les travaux de cette première convention se terminant au mois de janvier 2020, une nouvelle convention citoyenne portant sur un autre thème devrait être organisée au cours de l'année J'aurais aussi aimé savoir, monsieur le ministre, les suites qui pourront être données à cette première convention citoyenne, dont les débats semblent très suivis. Je conclus mon intervention sur les crédits de la Cour des comptes et des autres juridictions financières, qui restent quasiment stables hauteur de 220 millions d'euros, alors que la programmation pluriannuelle prévoyait une augmentation de près de 2 millions d'euros. Mes chers collègues, je vous invite à suivre l'avis de la commission des finances et à adopter les crédits de cette mission.

de l'État ; enfin, notre incompréhension après la décision de supprimer l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et nos inquiétudes sur les moyens de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). première remarque portera sur les crédits de personnel. Les effectifs progressent- c'est bien ! La structure d'emplois fait apparaître plus de cadres de haut niveau- c'était nécessaire Les contraintes salariales sont assouplies pour recruter des spécialistes dans les secteurs où les compétences disponibles sont rares et recherchées- c'était indispensable ! des coûts supplémentaires, les crédits de personnel de titre 2 sont en baisse de 17,6 %. Où est l'erreur ? Elle découle d'un jeu d'écriture entre le SGDSN et le ministère des armées. À partir de 2020, le programme 129 n'aura plus à rembourser les rémunérations des 255 militaires mis à disposition du SGDSN, de l'Anssi et du GIC. Ils resteront à la charge des armées, dont on sait que les crédits ont du mal à être consommés. Cet arrangement permet aux services du Premier ministre d'afficher un titre 2 en baisse et aux armées de consolider leurs crédits ! Jeu à somme nulle pour le budget de l'État, me direz-vous Certes, mais le titre 2 du programme 129 ne reflétera plus les « vraies » charges de personnel. Pour la représentation nationale, qui assure le contrôle des crédits, cette perte de lisibilité complique l'évaluation de la performance de ces administrations. Ces arrangements transforment petit à petit nos comptes publics en usine à gaz et nous éloignent d'une application rigoureuse de la LOLF. Je doute que cela améliore la performance publique deuxième remarque a trait à la cybersécurité. En 2018, l'Anssi a traité 78 événements de sécurité consécutifs à des attaques informatiques ayant touché des ministères.

Elles maintiennent nos administrations dans un état de vulnérabilité inquiétant, comme en témoigne le niveau effectif de conformité de systèmes d'information, qui fait l'objet d'un indicateur du programme 129. Certes, les plans ministériels de renforcement de la sécurité sont plus nombreux, mais ils restent sous-financés pour répondre aux enjeux. Nous sommes particulièrement inquiets pour le secteur de la santé et la protection des hôpitaux, qui se sont beaucoup digitalisés, mais sans réaliser tous les efforts de protection nécessaires, comme l'illustre l'attaque du centre hospitalier universitaire de Rouen,

Elle passe aussi par la reprise de la croissance des effectifs de l'Anssi, ralentie depuis deux ans, et par le desserrement de la contrainte salariale pour recruter des collaborateurs de bon niveau au prix du marché. À cet égard, le projet de loi de finances pour 2020 est satisfaisant et va dans le sens de nos recommandations. Sans portage politique majeur, sans moyens financiers significatifs et sans outils réglementaires plus coercitifs, il sera difficile de lutter contre une logique valorisant la multiplication des systèmes d'information et des applications numériques. également rompre avec la logique qui privilégie la baisse des coûts de fonctionnement ou de personnels des services de l'État, sans se préoccuper suffisamment de leur sécurité. Ma troisième remarque concerne la situation de l'IHEDN et de l'INHESJ. Il a été décidé de supprimer l'INHESJ à compter du 31 décembre 2020. Cet institut était pourtant devenu l'opérateur public de référence dans les domaines de la formation et de la recherche liées à la sécurité globale et à la justice un lieu par lequel sécurité et justice se renforcent des échanges avec le monde scientifique, grâce à des programmes de recherche de qualité ; un lieu de construction de référentiels communs pour des corps amenés à agir ensemble au quotidien, souvent en tension. commission des affaires étrangères ne comprend pas cette décision. La pérennité de l'IHEDN est assurée. C'est un soulagement ! Son nouveau plan stratégique constitue un net progrès, mais son modèle économique reste à construire. La stabilisation de sa trajectoire financière n'est donc toujours pas acquise. De surcroît, cet organisme devra absorber, seul, certaines charges mutualisées avec I'INHESJ et, peut-être, reprendre certaines formations dispensées. Avec quels moyens ? La commission, très attachée à cet institut, est en attente de réponses précises du Gouvernement. Globalement, l'économie pour le budget de l'État de cette opération de simplification reste à démontrer. Notre commission avait proposé de donner un avis favorable à l'adoption des crédits, mais c'était avant le coup de rabot infligé à l'Anssi et au GIC en deuxième délibération à l'Assemblée nationale ... Nous soutiendrons bien évidemment le rétablissement de ces crédits ! La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) chargée de l'élaboration et du pilotage de la politique gouvernementale dans ce domaine. Les résultats de cette politique sont encourageants. En 2019, le tabagisme continue à reculer dans notre pays, de même que la consommation globale de substances psychoactives par les plus jeunes, dont l'âge d'expérimentation recule, tandis que la consommation d'alcool se stabilise. Il convient toutefois de maintenir une vigilance particulière, outre sur l'alcool, sur certaines addictions sans substance, comme l'addiction aux écrans ou aux jeux vidéo, mais aussi sur certains excitants ou euphorisants très à la mode chez les jeunes, voire les très jeunes, comme le poppers ou le protoxyde d'azote. Les efforts de prévention doivent en outre être renforcés sur le cannabis, dont la consommation reste, en France, la plus élevée d'Europe, chez les adultes comme chez les jeunes. Le marché du cannabis aiguise les appétits d'industriels désireux de profiter des opportunités de légalisation ouvertes dans un nombre croissant de pays- récemment encore, au Luxembourg. Ne laissons pas sa banalisation s'imposer dans le débat public, car sa toxicité sur les jeunes cerveaux est avérée ! Pour relever ces défis, la Mildeca se trouve toutefois dans une situation triplement inconfortable. D'abord, ses crédits continuent de diminuer. Ils seront de 17,1 millions d'euros en 2020, soit une baisse de 2,3 % par rapport à l'année passée. Cette baisse correspond essentiellement à une diminution des effectifs de la mission et aux économies de loyer réalisées par son principal opérateur, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Reste que, entre 2012 et 2018, la baisse des crédits de cette mission avait déjà atteint 25 %. L'apport du fonds de concours « drogues », revenu à ses niveaux d'il y a dix ans, soit une vingtaine de millions d'euros, est quant à lui surtout un révélateur de la vigueur Ensuite, le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022, que la Mildeca est chargée de piloter, semble dépourvu de portage politique fort. Plusieurs fois reporté avant d'être annoncé au mois de décembre dernier, ce plan présente en définitive la luxuriance de plus de 200 mesures assez techniques- même si nous nous réjouissons qu'il tienne compte de certaines de nos recommandations.

à la recherche et de marketing social, fait planer sur la frêle Mildeca l'ombre assez menaçante de ses 120 millions d'euros ... En bref, le pilotage de cette politique gagnerait à être rationalisé, pour plus de cohérence, de lisibilité et d'efficacité. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dois d'abord informer le Sénat des conditions pour le moins singulières dans lesquelles j'ai été amené à rédiger mon rapport pour avis au nom de la commission des lois. En effet, malgré mes demandes réitérées, les services de l'Élysée ont refusé de recevoir le rapporteur que je suis ! Intolérable ! Or suis ! Intolérable ! Or cette audition avait lieu chaque année, sans que cela posât le moindre problème.

augmentent, passant de 106 780 000 euros à 110 516 000 euros. La dotation de l'État,

à moi, j'ai bientôt épuisé le temps de parole qui m'était imparti, mes chers collègues, pour vous parler de l'Élysée- je n'ai fait qu'effleurer le problème du Sénat, de l'Assemblée nationale, des chaînes parlementaires, du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de la République. Cela me permet une nouvelle fois, monsieur le président-

note que les juridictions administratives bénéficient d'une hausse de leur budget de 4,6 %. Toutefois, cette augmentation, qui représentera, et c'est important, 93 emplois nouveaux, est très inégalement répartie.

Celui-ci pourrait atteindre 53 % sur la période 2019-2020, avec près de 90 000 requêtes attendues, selon les estimations de l'Ofpra.

Pour le reste, comme l'année dernière, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel font figure des grands laissés-pour-compte de ce budget, avec seulement 34 emplois nouveaux. Ce renforcement des moyens humains est sans proportion avec l'augmentation du contentieux à laquelle sont confrontées les juridictions administratives, qui ont connu deux années consécutives de hausse sans précédent, en particulier dues aux contentieux des étrangers. L'augmentation des demandes d'asile se traduit en effet par un bond considérable du contentieux de l'éloignement et des référés-liberté.

collègues, compte tenu de l'effort conséquent envers la CNDA et du maintien à la hausse, même légère, des moyens accordés aux juridictions administratives et financières, Patrick Kanner estime juste que la commission des lois vous propose, conformément à son rapport

des droits et libertés », qui recouvre le budget des autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits et libertés. Je rappelle que les autorités administratives indépendantes sont des autorités administratives, dont il a été jugé indispensable qu'elles soient indépendantes de l'exécutif, de manière à mieux préserver les libertés

Monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le bric-à-brac que sont devenus les projets de loi de finances a cet avantage inattendu de permettre des rapprochements qui

l'idée saugrenue de fusionner la Miviludes, placée depuis sa création, en 2002, sous l'autorité du Premier ministre, avec le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation,

C'est à se demander quelles sont les véritables raisons de la mise à mort d'un organisme aussi essentiel, en ces temps de floraison des marchands de faux espoirs. à se demander si la Cour des comptes, qui a pris l'habitude de juger de tout, est, en l'occurrence, dans son rôle.

Les crédits de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », tels qu'ils figurent dans le projet de loi de finances pour 2020, sont maîtrisés, tout en finançant des priorités comme le numérique, la sécurité ou le renforcement des moyens de la CNIL et, dans une moindre mesure, les crédits du Défenseur des droits et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dans le projet de loi de finances initiale, ces crédits sont en hausse de 4,36 % en autorisations d'engagement et de 0,46 % en crédits de paiement par rapport à ceux qui ont été Les crédits du budget annexe « Publications officielles et information administrative » connaissent, quant à eux, une baisse significative. Cela s'explique par la réduction de personnels engagée depuis plusieurs années. viens au programme 129. Nous ne pouvons que nous féliciter des efforts continus en faveur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), chargée notamment de la protection des systèmes d'information des opérateurs essentiels à l'économie et à la société. Comme l'a rappelé M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères, ces enjeux sont cruciaux face aux cyberattaques, qui sont de plus en plus virulentes.

qui contribue à entretenir le lien de la Nation avec son armée, ne doit pas devenir la victime collatérale de cette diminution. En ces temps d'instabilité géopolitique et de menace diffuse, je crois plus que jamais utile pour notre pays le maintien de l'effort de formation et de sensibilisation aux enjeux de défense. Nous devons

nouvelles missions. La mission « Conseil et contrôle de l'État » verra ses crédits augmenter de 3,55 % en 2020. Cette hausse paraît justifiée par la nécessité de répondre à des contraintes spécifiques, dont certaines vont croissant.

Concernant le budget de la présidence de la République, qui cristallise toutes les attentions, surtout celle de notre collègue M. Sueur, la dotation demandée la dotation demandée pour l'année 2020 passe de 103 millions à 105,316 millions d'euros. Cette augmentation s'explique principalement par une mesure de périmètre périmètre recommandée par la Cour des comptes : la dotation inclura désormais les dépenses de fonctionnement et d'équipement de la sécurité de la présidence de la République. En conclusion,

de la présidence de la République et du Conseil constitutionnel. Je ne reviendrai pas sur la question de la Cour de justice de la République, qui survit et coûte cher, malgré le consensus incontestable en faveur de sa dissolution- cette question relève d'une réforme constitutionnelle. En 2020, les moyens de l'ensemble de ces institutions constitutionnelles s'établiront à plus de 994 millions d'euros, dont un peu plus de 841 millions pour le Parlement, soit environ 13 euros par Français et par an. C'est une transparence nécessaire que nous devons à nos concitoyens et dont il leur appartient de juger l'opportunité. Voilà le prix de la démocratie le prix de la démocratie ! La mise en oeuvre d'outils de démocratie directe et de participation citoyenne a également un coût. Pour le Conseil constitutionnel, le prolongement du suivi du référendum d'initiative partagée, organisé sur la seule question de l'avenir des régimes de gestion des Aéroports de Paris

Conseil et contrôle de l'État », s'élèvera à 4,2 millions d'euros. Il est vrai qu'à la différence des chambres parlementaires la ventilation du financement des outils de démocratie directe entre différents programmes et missions rend l'estimation de leur coût plus difficile pour le citoyen observateur. Ce n'est pas là le moindre des paradoxes. Cependant, ces données ne doivent pas être sous-estimées, à une époque de réflexion intense sur les évolutions institutionnelles de notre démocratie. La mission « Direction de l'action du Gouvernement » rassemble, quant à elle, les moyens mis à disposition du Gouvernement, placés sous l'autorité du Premier ministre. Elle concerne donc des services très variés, qui jouent souvent un rôle d'impulsion incontournable pour les politiques publiques conduites par l'État. Cette année, l'intégration du programme 333, « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées de l'État », au programme 307, « Administration territoriale de l'État », au sein de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » constitue la principale évolution,

Une fois décompté cet effet de périmètre, les moyens dévolus à l'action interministérielle augmentent donc de 4,4 % par rapport à 2019, avec d'importants contrastes sectoriels. Ainsi, comme l'ont souligné les rapporteurs spéciaux des deux assemblées, alors que certains services bénéficient d'un clair soutien financier, tel le service d'information du Gouvernement (SIG), dont le budget augmente de 1 million d'euros entre 2019 et 2020, d'autres ont subi des arbitrages plus sévères.

la souveraineté nationale face aux cybermenaces, comme l'ont noté plusieurs collègues. Plusieurs membres du groupe RDSE s'inquiètent en revanche

d'euros est attendu. Le groupe RDSE reste très attaché à l'action d'information du citoyen, menée avec beaucoup de sérieux par la Documentation française. Nous encourageons le Gouvernement à soutenir les efforts de renouvellement accomplis par les agents viens à la mission « Conseil et contrôle de l'action de l'État ». Je ne reviendrai pas sur la position du groupe RDSE sur les autorités administratives indépendantes, qui n'a pas varié depuis le rapport Mézard. En revanche, au regard du poids croissant du budget

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

aux victimes notent une augmentation des appels liés à ces églises. Monsieur le ministre, ne faudrait-il pas tenir compte des réunions en préfecture sur les dérives sectaires, qui font remonter des situations

de l'Église évangélique baptiste de toutes les nations (EBTN), a été mis en examen pour viols ; même chose pour un prêcheur de Colombes, accusé d'avoir violé plusieurs jeunes femmes. En 2018, à Draveil, une cinquantaine de plaintes ont été déposées par les adeptes d'une église évangélique pour une escroquerie avoisinant les 2 millions d'euros. Avec une stratégie d'expansion agressive, les églises évangéliques se sont implantées dans toute la France. Même si elles restent plus concentrées dans les villes et leur périphérie, elles s'installent aussi en zone rurale. Ces églises évangéliques jouent sur un réflexe communautaire- nous en parlons beaucoup sur d'autres sujets, pourquoi pas sur celui-ci -et visent des publics peu insérés socialement.

unique. L'année dernière, lors de l'examen de la mission « Pouvoirs publics », après avoir constaté la forte hausse du budget de la présidence de la République, inversement proportionnelle à la diète imposée aux Français et aux collectivités locales,

La crise des « gilets jaunes », sorte de cri lancé par la France d'en bas au Président de la République, aurait pu conduire à un peu de modération. Une fois encore, nous assistons à une augmentation des crédits alloués à la présidence de la République et à un épuisement programmé de ses réserves, au point qu'en 2021 celles-ci n'existeront plus. Si les pouvoirs publics sont soumis à un traitement budgétaire particulier, justifié par l'exigence d'autonomie financière liée à ces institutions, et déterminent eux-mêmes le montant des crédits dont ils ont besoin selon une procédure encadrée, la transparence, la baisse des dépenses publiques et l'exemplarité n'en sont pas moins indispensables, dans une période où les où les efforts imposés à nos concitoyens sont considérables. C'est ce qu'ont compris l'Assemblée nationale et le Sénat, avec des dotations reconduites à l'identique depuis 2012 ; leurs dépenses Comme le rappelle M. Bascher, rapporteur spécial de la mission « Pouvoirs publics », « avec l'inflation, cela signifie que [les assemblées parlementaires] ont perdu sur cette période l'équivalent d'une année de dotation par rapport à 2011. Les assemblées ont réalisé un effort important de maîtrise de leurs dépenses Le Parlement témoigne ainsi de sa volonté forte de participer pleinement à l'effort de redressement des comptes publics. Il eût été heureux que l'Élysée adopte la même rigueur et la même sagesse, la même transparence et la même modération.

Alors que l'État a imposé aux collectivités territoriales depuis deux ans, sous peine de forte pénalité financière, une contractualisation limitant à 1,2 % l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement, la présidence de la République s'autorise, quant à elle, une augmentation près de trois fois supérieure. peine rappeler, face à cette hausse de 3,5 %, le montant de la hausse des allocations familiales, de 0,3 % ou celle des pensions de retraites, comprise entre 0,3 % et 1 %, soit un montant bien inférieur à l'inflation. aurions pu espérer que cette forte hausse du budget de la présidence ait pour objectif louable l'entretien du patrimoine remarquable qui lui est confié et qui ne cesse de se dégrader. Alors que,

Il n'en reste pas moins que cette mission, même modeste, regroupe des budgets qui sont à nos yeux stratégiques, notamment en matière de sécurité numérique. Dans l'ensemble,

face à cette débudgétisation, qui entraîne une diminution des crédits un peu artificielle., nous sommes tout à fait satisfaits de la hausse des moyens en faveur de la sécurité numérique

Dans le même ordre d'idées, dans le programme 308, « Protection des droits et libertés », la CNIL obtient une dotation supplémentaire de 10 postes.

Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDSN, est évidemment l'un des fleurons de cet ensemble d'administrations. Il joue un rôle tout à fait essentiel pour la protection des intérêts nationaux et la coordination de tous les services associés

sénateurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier de vos interventions et à saluer le travail des rapporteurs, qui ont exposé les grandes lignes du budget sur lequel le Sénat doit se prononcer ce soir. Je m'efforcerai d'apporter des compléments d'information à ce qui a déjà été dit, ainsi que, dans la mesure du possible, des réponses à vos différentes interrogations.

D'ailleurs, les assemblées parlementaires font de même sur leur propre budget. Depuis plusieurs années, la Cour des comptes exhorte la présidence « à mener à bien les travaux liés à la conservation du patrimoine immobilier, au risque que celui-ci continue de se dégrader et que les coûts de sa restauration soient augmentés ». Il était grand temps de lancer un programme de travaux et la prise en charge d'une partie du financement de ce programme

Quant aux dépenses de fonctionnement, elles sont en très légère hausse en raison du « rebasage » que j'ai précédemment évoqué, pour un montant de 900 000 euros, des frais inhérents aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des militaires et policiers affectés à la direction de la sécurité de la présidence de la République. Tendanciellement, ces crédits de fonctionnement baissent grâce à un meilleur encadrement de la prise en charge des frais de déplacement, au contrôle de gestion,

attribuer un supplément exceptionnel de 785 000 euros de crédits lié au référendum d'initiative partagé sur la privatisation d'Aéroports de Paris. La Cour de justice de la République voit, quant à elle, ses crédits augmenter de 10 000 euros : il s'agit d'assurer le renouvellement de son parc informatique.

Face à un contentieux de l'asile particulièrement dynamique- si je puis dire -, la CNDA est apparue comme la juridiction dont l'augmentation des moyens devait être privilégiée. C'est la raison pour laquelle elle bénéficiera

à ce qu'il était en 2010. Pour ce qui est de l'interruption du remboursement des rémunérations des personnels mis à disposition du SGDSN, j'ai évidemment noté le scepticisme de MM. Canevet et Leconte ; s'y ajoutent les Cette décision fait suite à la volonté interministérielle d'associer le ministère des armées à la prise en charge de la coordination de la sécurité nationale et de la cyberdéfense. Je réponds aux Je réponds aux inquiétudes de MM. Canevet et Cadic au sujet de l'INHESJ. L'objectif est bien la reprise des formations et des activités par les ministères de la justice et de l'intérieur, dans le cadre d'un programme commun permettant de maintenir un haut niveau de coordination avec, le cas échéant, une session annuelle commune

des addictions au sens large, et ce dès le plus jeune âge. Comme Mme Harribey et M. Cadic, je me félicite de la hausse des moyens dévolus au GIC et à l'Anssi- à charge désormais à l'autorité politique de s'investir davantage, et au niveau adéquat, dans le pilotage interministériel de la sécurité des systèmes d'information.

La commission des finances émet un avis défavorable sur le sous-amendement et les trois amendements

supérieur de l'audiovisuel a été épargnée. Pour les autres autorités administratives indépendantes, les montants sont très limités : ils ne représentent pas plus de quelques dizaines de millions d'euros, ce qui nous paraît absorbable, compte tenu de ce qui s'est passé les années précédentes. Concernant le programme 129,

déjà créés en 2019. Par ailleurs, un décret de transfert sera examiné en gestion en 2020 afin de permettre à la HATVP d'examiner les saisines obligatoires que devront formuler auprès d'elle les agents publics en cas de départ vers le secteur privé ou de cumul d'activités, une compétence reprise à la Commission de déontologie de la fonction publique, en application de la loi du 6 août 2019 Les crédits hors titre 2 de la HATVP augmentent, par ailleurs, de 1 million d'euros en autorisations d'engagement et de 0,2 million d'euros en crédits de paiement. Cette augmentation résulte principalement de l'extension de l'implantation de cette autorité dans les locaux loués par le Conseil d'État.

2018. Hors correction technique liée au transfert du titre 3 vers le titre 2 des personnels de droit privé mis à disposition par des organismes de sécurité sociale, leurs moyens, hors titre 2, sont bien en progression nette. En conséquence, il nous semble que les moyens proposés sont conformes aux besoins budgétaires du Défenseur des droits. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet

dont l'Anssi dispose pour assurer la cybersécurité de l'ensemble du pays soit maintenu, que la trajectoire

Le SIG a été réorganisé en 2019, pour répondre aux nouvelles missions de transformation digitale de la communication gouvernementale, qui lui ont été confiées par la circulaire du 27 mars 2018. La structure favorise désormais une gestion intégrée des projets de communication, depuis l'analyse de l'opinion, la définition de la stratégie de communication, jusqu'à la diffusion des campagnes et l'analyse de leur impact sur l'audience. La parole